M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 27 juin dernier portant convocation du Parlement en session extraordinaire. Acte est donné de cette communication. Ce décret, qui vous a été adressé, mes chers collègues, a été publié sur le site internet du Sénat. En conséquence, la session extraordinaire est ouverte. M. Dominique Watrin a fait connaître à la présidence qu'il se démettait de son mandat de sénateur du Pas-de-Calais, à compter du 30 juin 2018, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par Mme Cathy Apourceau-Poly, dont le mandat de sénatrice du Pas-de-Calais a commencé le 1 juillet, à En application de l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, une communication de laquelle il résulte que, à la suite des opérations électorales du dimanche 1 juillet 2018, M. Vincent Segouin a été proclamé sénateur de l'Orne. Son mandat a débuté lundi 2 juillet, à zéro heure. Au nom du Sénat tout entier, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

En effet, l'étude d'impact souligne que ces pratiques auraient pour effet d'encourager l'acquisition et l'utilisation de plus de produits que strictement nécessaire pour répondre aux besoins de leurs exploitations. marquait une avancée importante, car, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nier que l'utilisation abusive des pesticides pose un problème de santé publique. Pour les agriculteurs et leurs proches, pour les riverains et les consommateurs, l'utilisation de ces produits se traduit par une augmentation des risques d'apparition de maladies graves, de complications dans le développement des foetus et des très jeunes enfants exposés, sans parler des effets cumulés sur la santé de l'ensemble des expositions aux PPP, qu'on appelle « effet cocktail Dès lors, nous nous interrogeons sur la position du Sénat, qui semble céder à des intérêts purement économiques de court terme, face aux enjeux immenses que l'utilisation des PPP représente en matière de santé et d'environnement. C'est pourquoi nous proposons de rétablir l'article 14 dans sa rédaction initiale. Il est impératif de réduire l'utilisation des pesticides, et ce dès maintenant. La

pour les agriculteurs, dont les maladies professionnelles se développent, ainsi que pour l'environnement. De plus en plus d'études démontrent l'étendue de leur effet. En parallèle, malgré les sommes d'argent public importantes consommées par les plans Écophyto successifs, la quantité de pesticides utilisés continue d'augmenter. Accepter des pratiques commerciales poussant à la consommation, comme des remises et des rabais, paraît ainsi complètement inapproprié au regard de la volonté publique politique nationale.

n° 551 rectifié. Il s'agit d'un amendement de rétablissement d'un article, supprimé en commission, qui visait à interdire certaines pratiques commerciales se déroulant traditionnellement à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques : les « 3 R »- remises, rabais, ristournes -, les différenciations des conditions de vente en fonction des acheteurs, la remise d'unités gratuites ou des pratiques équivalentes. Puisque nous considérons que les produits phytopharmaceutiques ne sont pas des produits comme les autres, Joël Labbé vient encore de le rappeler, en raison de leur dangerosité potentielle et avérée, il nous semble nécessaire d'adopter des comportements visant à réduire leur usage et, surtout, de ne pas les assimiler à des produits agricoles classiques qui ne présentent pas de danger pour la santé des utilisateurs ou des consommateurs finaux. Je rappelle que la mission d'information sur les pesticides que nous avions menée ici même en 2012, dont j'étais la rapporteur et Sophie Primas la présidente, a

monsieur le ministre, pour les produits phytopharmaceutiques, telle qu'elle est issue des débats de l'Assemblée nationale. L'article 14 a pour objectif d'éviter toute incitation commerciale à utiliser des produits phytosanitaires de manière inappropriée, alors que, pour des raisons de santé publique et de protection de l'environnement, il est essentiel de diminuer l'utilisation conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans son plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides. Cet article est analogue à l'article introduit dans le code de la santé publique par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a interdit les remises, rabais et ristournes à l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques et qui a grandement contribué au succès du plan Écoantibio dont j'ai fait état ici même la semaine passée.

d'autant que, sur ce point, la commission a estimé, au même titre que le Conseil d'État, que, en l'absence d'étude mesurant l'impact de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques pour le monde agricole,

Or le caractère transposable de cette mesure n'est pas convaincant. En tout état de cause, il est assez douteux ! L'usage de médicaments diffère totalement de celui des produits phytopharmaceutiques. En outre, les professionnels de l'élevage ont indiqué à plusieurs reprises que la tendance à la baisse de la consommation était liée uniquement à cet encadrement des pratiques commerciales, mais bien davantage à une adaptation des pratiques des agriculteurs eux-mêmes et à la mise en place d'une véritable politique de prévention des maladies dans les élevages.

mesure semble traduire l'idée que, si l'agriculteur utilise davantage de produits, c'est parce qu'il les achète en promotion. Je crois qu'il faut bien réaffirmer que les agriculteurs sont les premières victimes de ces produits et que c'est non pas la promotion qui fait l'usage, mais bien la nécessité et l'absence d'alternative de traitement. Dès lors, la commission est défavorable à l'ensemble des amendements.

c'est une méconnaissance totale des efforts menés par toute une profession pour utiliser les meilleures techniques, afin de limiter au maximum leur emploi. Informatique embarquée, bas dosage, Certiphyto ... Tous ces mots riment avec technicité, responsabilité et application. c'est une réelle injustice. Comment expliquer que seuls les agriculteurs seraient punis, alors que, partout ailleurs, les rabais, remises et ristournes font partie intégrante des négociations commerciales et sont les éléments clés d'une diminution des charges que toute entreprise bien gérée se doit de faire ? Comment peut-on maintenir que cette mesure est une bonne mesure, compte tenu de l'actualité et des ristournes accordées durant la campagne du candidat Macron ? Comment le Gouvernement pourra-t-il maintenir devant tous les agriculteurs de France qu'il rencontrera dans les jours à venir que cette mesure n'est pas le nouveau produit d'une politique du « deux poids, deux mesures » ? Interdire 1 % de remise aux paysans, alors que notre Président de la République a bénéficié de remises pouvant atteindre 60 % à 70 %, est tout simplement indécent.

favorisant l'utilisation des biocontrôles et en faisant en sorte que, dans une stratégie bien définie avec les agriculteurs, conformément à ce que ceux-ci souhaitent à travers le projet de « contrat de solutions

Pourquoi ne pas continuer dans la même voie ? Nous avons vu les dangers de la politisation et de la médiatisation à outrance de certains dossiers, comme celui du glyphosate.

Nous avons également vu les dangers et les problèmes créés par la surtransposition de la réglementation européenne. Ce débat nous offre donc une excellente occasion de mettre en adéquation nos paroles et nos actions.

C'est la raison pour laquelle je reste particulièrement ferme- et serein -sur cet amendement.

domaine. La société allemande est en train de bouger, tout comme bouge la société française. Les consommateurs, nos concitoyens, nous réclament des comptes sur ces sujets. Pour autant, nous ne devons pas faire les choses n'importe comment. Nous devons accompagner cette transition. Vous aurez remarqué que je ne fais pas partie de ceux qui prennent pour postulat de départ d'interdire les choses de manière brutale. Au contraire, je souhaite utiliser le temps

phytopharmaceutiques concernant notamment les conditions d'étiquetage qu'ils doivent respecter et l'interdiction de vente en libre-service de certains produits aux particuliers. Le contrôle des produits phytopharmaceutiques est notamment réalisé par les agents de la concurrence,

parole est à Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement d'appel vise à demander au Gouvernement de s'engager auprès de ses partenaires de l'Union européenne pour demander la création d'un fonds interagences sanitaires au niveau européen aurait pour but de financer des études et travaux de recherche sur les risques sanitaires et environnementaux insuffisamment documentés ou controversés. Ce dispositif permettrait, d'une part, de répondre à des situations de crise se caractérisant par des controverses scientifiques ou sociétales et, d'autre part, d'agir de façon

dans le cadre du plan de sortie des produits phytosanitaires que j'ai présenté le 25 avril dernier avec trois de mes collègues. Nous avons salué la position de la Commission européenne, qui propose aussi la création d'un tel mécanisme. La Commission a accepté de mener des études

pour certaines catégories de produits biocides qui seront définies par décret. Il s'agit de produits de la vie courante- désinfectants ménagers, produits de protection du bois, insecticides -ayant un intérêt sanitaire qui visent à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles par une action chimique ou biologique. Dans un contexte de recrudescence des nuisibles, en France métropolitaine comme dans les départements et collectivités d'outre-mer, le maintien d'un accès raisonnable aux produits biocides constitue un enjeu de santé publique majeur. L'utilisation et la mise sur le marché de ces produits étant d'ores et déjà régies par le règlement européen n° 528/2012, l'article 14 constitue une surtransposition injustifiée susceptible de créer une distorsion réglementaire vis-à-vis des autres États membres.

Ce sujet soulève de véritables problèmes sanitaires : le contrôle des nuisibles est un enjeu de santé publique et l'accès à ces produits, y compris par les utilisateurs non professionnels, est nécessaire.

des perturbateurs endocriniens. Pour ces raisons, je suis défavorable à la suppression de l'article 14 La

le rappelle, un premier volet de cet article visait à transposer aux produits biocides les interdictions de pratiques commerciales prévues par l'article 14 pour les produits phytopharmaceutiques. Cette disposition a été supprimée par la commission des affaires économiques, par parallélisme avec la suppression de l'article 14. L'article 14 comprenait deux autres dispositions, qui ont été maintenues : d'une part, une interdiction de la vente en libre-service aux particuliers de certaines catégories de produits biocides ; d'autre part, une interdiction de la publicité commerciale pour certains de ces produits biocides. Ces dispositions tendaient donc à transposer à certaines catégories de produits biocides des dispositions appliquées depuis plusieurs années aux produits phytopharmaceutiques. Favorable à cette évolution, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a proposé d'apporter des précisions sur les obligations d'information à la charge des distributeurs. Nous avons par ailleurs prévu que le décret identifiant ces produits devra définir le calendrier du programme de retrait dans les lieux de vente pour donner de la prévisibilité aux entreprises concernées. Ces modifications, qui avaient été acceptées par la commission des affaires économiques lors de l'élaboration du texte de la commission, ont permis d'améliorer la rédaction de l'article 14 Compte tenu de l'avis favorable émis à l'instant sur ces amendements de suppression, je souhaite rappeler que cet article ne vise que certaines catégories de produits identifiés en raison de leurs risques sanitaires et environnementaux. En outre, il ne tend aucunement à interdire l'utilisation des produits concernés. Je souligne enfin que de nombreuses substances actives utilisées dans les produits phytosanitaires se retrouvent également dans les produits biocides. Si l'on souhaite réduire l'exposition quotidienne de la population aux substances chimiques et mieux protéger l'environnement, il est pertinent d'encadrer la distribution et la publicité des biocides en s'inspirant de ce qui fonctionne bien pour les produits phytosanitaires. La commission du développement durable est donc attachée au maintien de ces deux dispositions, telles qu'elles résultent des travaux de la commission.

un agriculteur, un consommateur ou un riverain d'une parcelle traitée se trouve en contact avec une variété de substances, dont les effets peuvent se combiner pour représenter une toxicité imprévisible et potentiellement supérieure à celle de chaque molécule prise séparément. L'évaluation des risques est aujourd'hui fondée sur des méthodes qui n'intègrent pas, sauf cas spécifiques, les effets des mélanges de molécules,

L'évaluation des risques doit désormais aussi prendre en compte la réalité des effets cocktail et de leur impact sur la santé publique, notamment pour les plus vulnérables, comme les femmes enceintes et les jeunes enfants. L'ANSES a commencé ce travail, mais il reste encore marginal. Peu d'informations sont disponibles, alors qu'il s'agit là d'une mission essentielle.

Il ne s'agit pas, mon cher collègue, de sous-estimer le risque de ces effets, qui sont encore à découvrir. Vous l'avez dit, l'ANSES a commencé un travail sur le sujet, son projet Périclès, qui vise à développer une méthode pour déterminer les mélanges les plus fréquents auxquels la population est exposée dans son alimentation

dans la prise en compte des effets cocktail des produits phytopharmaceutiques sur la santé de l'homme. Les études de l'INSERM et de l'ANSES montrent, dans un certain nombre de situations, des risques potentiels pour la santé humaine liés à ces effets cocktail ou « effets mélange ». Comme le précisait le rapport d'information de 2012, le danger de cet effet cocktail est le suivant : « Différentes substances peuvent avoir un effet additionnel, antagoniste, voire synergique, à savoir ne pas produire d'effet notable individuellement, mais produire un effet important lorsqu'elles sont administrées, de manière combinée, à des doses sans effet. » Or « les procédés d'évaluation des risques en place actuellement ne permettent aucunement de mesurer ces effets cocktail potentiels Nous estimons que cette situation ne peut perdurer. La prise en compte des effets cocktail, notamment dans le cadre de l'évaluation des PPP, doit devenir demain une priorité. C'est pourquoi, afin qu'un travail clair soit engagé dans ce domaine, nous souhaitons que le Gouvernement nous remette un rapport dressant un bilan de la recherche dans ce domaine, qui nous servira de base à une modification de notre

en légalisant, sans passage par l'ANSES comme c'est prévu aujourd'hui, l'usage biostimulant de toutes les plantes ou parties de plantes qui sont consommées dans l'alimentation humaine. La nouvelle rédaction modifie complètement l'esprit de l'article, en réintroduisant une obligation d'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

biodégradables et utilisées à faible dose. Parce qu'elles sont à base de molécules naturelles, elles se dégradent facilement. Actuellement, Les autres, soumises à évaluation, sont autorisées par une procédure nationale en dehors du cadre de la réglementation des pesticides. Or cette évaluation est inutile pour cette catégorie de plantes, à savoir les plantes autorisées

L'article 14 adopté par l'Assemblée nationale mettait donc en application l'avis donné au Gouvernement par ses propres experts de la Comtox, chargée de l'évaluation, qui a été transférée à l'AFSSA, puis à l'ANSES. Pourquoi prévoir une évaluation de l'ANSES pour des substances déjà évaluées ? Je tiens à votre disposition cette évaluation, pour quiconque souhaiterait la consulter ! La procédure simplifiée existant à l'heure actuelle n'est absolument pas opérante. Ces PNPP sont du domaine public. Aujourd'hui, l'ANSES demande, pour des produits pour lesquels aucune entreprise ne peut capter de la valeur, de faire des dossiers quasi identiques à ceux qui sont présentés par des producteurs de produits phytosanitaires. Aucun acteur n'a les moyens de le faire, et la situation reste bloquée. Je suis saisi

par notre commission ne change rien au droit actuel. Les termes « évaluation simplifiée » n'impliquent aucun changement, puisque les modalités sont toujours fixées par voie réglementaire. Or ce cadre réglementaire n'a jusqu'à présent autorisé que des plantes médicinales. Je rappelle que les produits médicinales. Je rappelle que les produits phytopharmaceutiques ont des conséquences graves pour les sols, l'air et l'eau. À l'heure où la valeur nutritionnelle de nos aliments diminue à force d'utiliser ces produits, il est essentiel d'en limiter l'usage pour la viabilité future de nos sols.

adopté par l'Assemblée nationale. La modification apportée par le Sénat n'est pas de nature à garantir la clarification et la simplification nécessaires pour l'utilisation des

Il tend à autoriser l'usage de toutes les plantes ou parties de plantes consommables dans l'alimentation humaine comme biostimulants. Il s'agit de promouvoir des alternatives naturelles aux pesticides, aux pesticides, moins coûteuses et moins dangereuses pour les producteurs. Je l'ai rappelé, ces solutions ont déjà été évaluées en 2001.

l'établissement de procédures spécifiques et de visas par l'ANSES, qui est par ailleurs débordée, je l'ai dit. Si ces plantes peuvent être consommées dans l'alimentation humaine, c'est bien qu'elles ne présentent pas de risques particuliers.

justifier l'interdiction de ce qui est utilisé sous nos fenêtres ? Pourquoi maintenir dans l'illégalité des agriculteurs et des jardiniers, mais aussi de petites entreprises artisanales dont les pratiques sont vertueuses, alors que, au même moment, on retire régulièrement des pesticides du marché,

ailleurs, j'ai été alerté sur l'importance de cette problématique dans nos outre-mer. Nos départements et régions d'outre-mer font face à une situation critique, 70 % des productions locales n'étant pas couvertes par la législation actuelle.

évaluation simplifiée par l'ANSES permettra d'émettre des recommandations concernant l'utilisation plus rapidement et plus facilement, qui préciseront les doses à utiliser. Tous ces paramètres sont nécessaires avant une commercialisation. Cette évaluation sera donc plus courte et simplifiée. Il s'agit bien d'une disposition simplificatrice,

chimiques. Les grosses sociétés, celles qu'on appelle les firmes, que j'accuse régulièrement, s'efforcent d'acheter ces petites entreprises pour prendre leur savoir-faire.

L'objectif de cet ajout est de prévoir par voie réglementaire une procédure adaptée à ces substances en vue de faciliter leur utilisation comme alternative aux produits conventionnels, sans pour autant les soustraire à toute évaluation préalable. Une telle modification est cohérente avec les recommandations faites par l'ANSES dans son avis technique de mars 2018 sur les critères d'évaluation des substances naturelles à usage biostimulant.

? Je le reconnais volontiers, les parties consommables des plantes présentent moins de risques, notamment pour la santé humaine. Comme l'ANSES l'indique dans son avis publié en mars dernier

Le texte est également en recul concernant la séparation de la vente et du conseil. Pourtant, les agriculteurs ont tout intérêt à avoir un conseil indépendant. Ils sont même 70 % à le réclamer. Un rapport de l'ANSES souligne un risque de conflit d'intérêts en cas de non-séparation de la vente et du conseil. Ces mesures vont à contre-courant du sens de l'histoire. Il nous faut préparer l'ère de l'après-pesticide. On doit pouvoir se passer de ces produits dangereux pour la santé, en tout premier lieu la santé des agriculteurs. Or les systèmes d'évaluation des molécules laissent à désirer. Peu transparents, ils se basent sur des dossiers fournis par les firmes de l'agrochimie. L'affaire des « Monsanto papers » l'a montré : ces études sont volontairement biaisées De plus, l'étude des effets chroniques se base uniquement sur la substance active, et non sur le produit avec ses coformulants, alors que ceux-ci se révèlent parfois plus toxiques que la substance active seule. Dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché, il est considéré que tous les agriculteurs portent des équipements de protection. Nous savons que c'est faux. Et le chiffre selon lequel les équipements de protection réduisent de 90 % les risques d'utilisation des produits n'est absolument pas démontré ; il semble même invalidé par un rapport de l'ANSES,

Il permet de déroger à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques dans les espaces verts- c'est le dispositif « zéro phyto » -ou par des non professionnels dès lors qu'il s'agit de lutter contre tout danger sanitaire. Je rappelle que le droit en vigueur n'applique pas ces interdictions aux produits de biocontrôle, aux produits à faible risque et aux produits utilisés en agriculture biologique. Surtout, le code rural et de la pêche maritime prévoit déjà des dérogations à l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques conventionnels lorsque seuls ces produits permettent de lutter contre les organismes nuisibles définis par voie réglementaire comme « danger sanitaire majeur ». Si cela est nécessaire, le droit en vigueur permet au ministre de l'agriculture de modifier la classification des dangers sanitaires pour autoriser l'utilisation de produits conventionnels contre de nouvelles menaces., menaces., en visant l'ensemble des dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment ceux d'importance mineure, de troisième catégorie, l'article 14 AA constitue une remise en cause excessivement large de dispositions importantes pour limiter l'exposition de la population aux produits phytopharmaceutiques.

autorisés lorsque l'application de produits de biocontrôle ou de préparations naturelles peu préoccupantes ne permet pas de lutter contre une maladie végétale connue. Cet article revient sur la loi adoptée en 2014, qui était pourtant véritablement consensuelle.

pour les cas extrêmes. Généraliser la possibilité de recours à la chimie en dehors des cas déjà prévus viderait la loi de tout sens. L'article 14 AA constitue donc un retour en arrière injustifié,

proposent des solutions très efficaces et alternatives à la chimie. Certaines sont appliquées dans les jardins prestigieux et patrimoniaux. Cet article est également injustifié du point de vue économique. La loi de 2014 a permis à de nombreuses TPE et PME françaises avec lesquelles je suis régulièrement en contact de développer des produits alternatifs aux pesticides. Elle est bénéfique pour l'emploi, puisqu'elle permet de créer des emplois locaux nouveaux et des innovations très intéressantes pour notre économie locale. Elle est évidemment bénéfique pour la santé des travailleurs : comment justifier de continuer à exposer les travailleurs d'espaces verts à des risques professionnels alors que des produits alternatifs existent ? En outre, l'article est injustifié du point de vue de la biodiversité. Au regard de la situation actuelle, nous avançons trop lentement. Si nous nous permettons en plus de voter des reculs sur les protections existantes appliquées sans difficulté sur le terrain, c'est que nous sommes

par rapport aux dispositions de la loi du 6 février 2014, dite loi Labbé, qui avait été modifiée par la loi d'août 2015, dite loi Potier. L'article semble considérer que seuls les produits phytopharmaceutiques dits conventionnels permettent de lutter contre les dangers sanitaires méconnaissant les principes de la lutte intégrée. Celle-ci privilégie les méthodes non chimiques, la prophylaxie, la surveillance, la prévention, le choix des espèces, les variétés.

Le scrutin est ouvert.

L'utilisation par les agriculteurs de mélanges de semences pour effectuer leurs semis est une pratique en constante augmentation, notamment en agriculture biologique. L'intérêt agronomique de l'utilisation de mélanges de semences consiste principalement à diminuer l'utilisation d'intrants par les agriculteurs, en sélectionnant des variétés complémentaires dans la résistance aux maladies. En dépit de l'intérêt évident de cette pratique, de nombreux freins en pénalisent le développement. Sur le plan du droit, la directive européenne 66/402 du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales, précise ainsi que les États « admettent que des semences d'une espèce de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés ». Cette directive n'a toutefois pas été transposée la réglementation française maintient le principe de l'interdiction de la commercialisation de mélanges de semences. C'est la raison pour laquelle, afin de lever ce frein et pour offrir une opportunité supplémentaire à nos agriculteurs, dans un contexte de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, il est proposé, au travers de cet amendement, d'inscrire explicitement dans la loi la possibilité de commercialiser des semences sous forme de mélanges de variétés. Quel

Actuellement, l'échange de semences doit respecter une procédure complexe, qui oblige à enregistrer la variété de semences au catalogue. Cet impératif ne fait pas la différence entre un échange à but commercial et un autre. Nous proposons donc, en accord avec les règlements européens et français, d'opérer une simplification quant aux règles d'échange de semences à but non commercial. Tandis que nous travaillons à réduire l'usage de produits phytopharmaceutiques, que nous cultivons de plus en plus de produits biologiques et agroécologiques et que nous opérons une transition vers une consommation durable et fondée sur les circuits courts, il est nécessaire de permettre une adaptation des cultures en fonction des régions. Les dernières décennies de standardisation des espèces de fruits et légumes nous ont fait perdre une pluralité qui témoignait des diversités régionales. Aujourd'hui, grâce à des variétés de semences anciennes, des paysans réussissent l'exploit de faire pousser en montagne des variétés rares de tomates, et ce sans intrants chimiques. Ainsi, l'usage des semences paysannes est l'occasion de diversifier l'agriculture, mais aussi de faire revivre les particularités de nos régions. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cette mesure pour la biodiversité de nos territoires. Quel ? Cet amendement reprend la rédaction du code rural. Il apparaît plus simple de vérifier que l'utilisateur n'est pas professionnel plutôt que de contrôler que l'utilisateur, quel qu'il soit, envisage ou non de suivre une exploitation commerciale de la semence. En outre, la rédaction proposée pourrait être interprétée de façon extensive et concerner plus que les jardiniers amateurs aujourd'hui visés par la dérogation. L'avis est donc défavorable. ? La modification ne change pas les difficultés que soulève pour le Gouvernement l'extension prévue à cet article de l'exemption d'inscription au catalogue des variétés cédées à titre onéreux à des utilisateurs professionnels. L'article, même ainsi rédigé, n'est pas conforme au droit européen et conduit à limiter l'information des utilisateurs

L'objet de l'amendement est d'organiser un recensement des variétés non enregistrées au catalogue et cédées à titre onéreux au travers d'une simple déclaration préalable dématérialisée qui pourrait contenir une dénomination et une description de la semence. Cela permettra d'avoir une vision exhaustive des variétés anciennes utilisées par les jardiniers amateurs et non inscrites au catalogue, sans pour autant ajouter une charge trop lourde à ces derniers.

Les directives concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, applicable à la quasi-totalité des variétés de semences, prévoient, à leur article 3, que « chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire ». Les dispositions de l'article 14 A en ce qu'elles exonèrent d'inscription au catalogue la cession à titre onéreux de semences ne sont pas conformes aux règles européennes. La cour d'appel de Nancy a confirmé cette interprétation dans un arrêt rendu en 2014. La directive de 2009 prévoit, par exception et pour les légumes, des critères d'admission allégés pour les variétés de conservation ou sans valeur intrinsèque, adaptées à des conditions géographiques particulières. Elle permet également d'exonérer de la procédure d'examen officiel les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières lorsque les informations détenues sont suffisantes. Dans ce contexte, et afin de faciliter encore la mise à disposition de ces semences tout en assurant une information minimale des jardiniers amateurs et le respect des dispositions européennes, il est proposé une procédure d'enregistrement des variétés qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 23 de la directive de 2009. Cette disposition devrait permettre de satisfaire la demande d'une réglementation adaptée et allégée pour la vente aux jardiniers amateurs et aux utilisateurs, mais aussi pour des pour des raisons de droit de concurrence. Enfin, afin de prévenir les risques sanitaires ou l'introduction d'espèces invasives sur le territoire national, il importe que le respect des règles sanitaires et leur contrôle s'appliquent aussi à l'étape de la commercialisation.

la publicité pour les produits phytosanitaires. Je crois qu'il a été question d'un parallélisme des formes entre l'alcool, le tabac et les produits phytosanitaires.

parole est à M. Henri Cabanel. Des agriculteurs, pour la plupart regroupés en réseaux, élaborent des stratégies locales et des expérimentations qui permettent de chercher, de développer et de promouvoir des modes de production durables, adaptés aux cultures et aux territoires divers dans lesquels ils s'inscrivent. Ces recherches ne sont pas nécessairement organisées ni produites par des organismes de recherche compétents. Elles n'en sont pas moins précieuses. Cet amendement vise à reconnaître l'engagement de ces agriculteurs attachés à sauvegarder le bien commun et à faire vivre un savoir-faire. Cette stratégie nationale doit en effet s'accompagner d'une collecte de bonnes pratiques locales qui ont déjà été testées sur le terrain ou peuvent l'être par des réseaux de paysans expérimentateurs, soucieux de faire évoluer les modes de production. Ceux-ci peuvent être considérés comme des partenaires à part entière. Ces « paysans chercheurs » ne sont pas à ce jour éligibles au crédit d'impôt recherche, puisqu'ils ne consacrent pas l'exclusivité de leur travail à la recherche. À ce titre, cet amendement vise également à proposer la création d'un crédit d'impôt recherche agricole qui pourrait être adapté à ces expérimentations

Cet amendement était initialement un amendement de repli, mais l'article 40 est malheureusement passé par là. Je le précise, car je ne voudrais pas que vous croyiez que je vous propose ici un énième rapport Dans notre amendement initial, nous proposions la mise en place d'un dispositif de soutien et d'accompagnement spécifique pour les entreprises s'engageant dans le développement du biocontrôle. En effet, aujourd'hui, beaucoup d'innovations en matière de biocontrôle sont le fait de start-up, de PME et de TPE. Or, souvent, ces dernières ne disposent pas des moyens suffisants pour produire des données nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché. L'ANSES, avec qui j'ai travaillé cet amendement, regrette ainsi de ne pas être en mesure d'instruire des dossiers ne comportant pas les données sur l'efficacité et la sécurité des produits exigées par la réglementation européenne. Cette situation est un frein évident au développement de ces techniques alternatives aux produits phytosanitaires classiques. C'est pourquoi nous estimons nécessaire, voire urgent, de permettre à ces entreprises de bénéficier des dispositifs de soutien à l'innovation. Malheureusement, comme je le disais en préambule, notre amendement a été retoqué au titre de l'article 40. Pour autant, je souhaiterais, mes chers collègues, ne pas écarter ce sujet central, qui s'inscrit totalement dans la démarche agroécologique et la transition de nos modèles de production. Je vous propose donc que le Gouvernement pose la première pierre de cet édifice en remettant un rapport au Parlement sur la mise en place d'un dispositif de soutien et d'accompagnement spécifique pour les entreprises s'engageant dans le développement du biocontrôle.

de compétitivité mis en place par la loi de finances pour 2005, à instituer des pôles de recherche et de développement de produits de biocontrôle. Si la France veut réellement amorcer un virage en matière de réduction de produits phytopharmaceutiques, notamment pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés dans le cadre du plan Écophyto, elle doit se doter d'une filière de recherche et de développement de produits alternatifs Les produits de biocontrôle sont l'un des leviers à activer. Or, comme je l'ai souligné, beaucoup d'innovations en matière de biocontrôle sont le fait de PME, de TPE et de start-up, qui rencontrent des difficultés pour mener à bien leur projet. C'est pourquoi le présent amendement vise à mettre en place des pôles de recherche et de développement du biocontrôle du biocontrôle afin de réunir dans une même entité toutes les forces en présence sur un territoire pour mettre en oeuvre des dispositifs de substitution aux produits conventionnels. Là aussi, cette position s'intègre parfaitement dans la transition agroécologique que nous appelons de nos voeux.

De même, un réseau de chercheurs sur le biocontrôle, le « réseau EMBA », s'est créé en 2014 associant des chercheurs de l'INRA et des industriels pour partager leurs travaux sur le biocontrôle.

par le groupe socialiste et adoptée à l'unanimité par la Haute Assemblée le 1 février 2018. Ce fonds vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits. L'amendement n° 559 rectifié concerne tous les malades, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Il vise à reprendre l'intégralité de la proposition de loi adoptée au Sénat en février. L'amendement n° 560 rectifié est une forme de « repli » dans le sens où il prévoit, dans un premier temps, de restreindre le champ de ce fonds aux maladies reconnues professionnellement. Notre proposition est totalement en adéquation avec les conclusions d'un rapport de janvier 2018 publié et des espaces ruraux. Ce fonds permettra d'accompagner les victimes qui souffrent de maladies liées à l'utilisation de ces produits en facilitant leurs démarches, en leur offrant un cadre global pour une plus grande égalité et en les indemnisant en réparation de l'intégralité du préjudice subi. Il permettra également de mieux identifier toutes les victimes, puisqu'on estime que seulement un malade sur dix est actuellement suivi pour cette raison. Monsieur le ministre, mardi, lors de la discussion générale au cours de vous avez déclaré que « nous avançons » sur la question du fonds d'indemnisation. Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas, et le moment est enfin venu d'accorder aux victimes la juste compensation qu'elles doivent recevoir.

Primas en 2012 sur ces sujets. Un rapport des inspections générales, qui a été remis en février 2018, préconise d'améliorer la réparation dans le cadre du régime accidents du travail et maladies professionnelles. C'est sur ce point que nous avançons en particulier.

les décisions de reconnaissance qui ne relèvent pas des tableaux de reconnaissance par les comités régionaux. Ce sera fait d'ici à la fin de l'année 2018. Nous avons voulu entamer une concertation pour améliorer l'indemnisation des exploitants agricoles dont le niveau d'indemnisation est moindre aujourd'hui que pour les salariés agricoles. En résumé, nous souhaitons améliorer améliorer le système d'indemnisation pour les victimes des produits phytopharmaceutiques par le dispositif qui existe aujourd'hui pour les maladies professionnelles. Par ailleurs, nous souhaitons répondre aux besoins

des produits phytopharmaceutiques puissent être mieux indemnisées, mieux traitées et qu'elles puissent faire valoir leurs intérêts Votre proposition initiale a été modifiée pour la limiter aux seules personnes dont la maladie a été reconnue comme maladie professionnelle consécutive à l'exposition aux produits phytopharmaceutiques. Vous avez ainsi pris en considération

les personnes victimes de maladies professionnelles liées à d'autres causes seraient indemnisées de manière moins favorable. En outre, certaines de ces maladies peuvent être causées par l'exposition à d'autres risques chimiques que des produits phytopharmaceutiques. Un tel dispositif, qui viserait à la réparation intégrale, exonérerait

et les industriels bénéficieraient, de fait, d'une décharge de responsabilité individuelle contre une prise en charge mutualisée du risque, sachant que les contributions qu'ils peuvent apporter concourent

dans le sens d'une meilleure reconnaissance et d'une meilleure traçabilité pour celles et ceux qui sont atteints par des maladies ou pathologies liées à l'utilisation ou à l'exposition à des produits phytosanitaires. Avec Mme

Il faut bien sûr agir prioritairement à la source du problème dans une logique préventive, en réduisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et l'exposition à ces produits à la fois pour leurs utilisateurs et la population ; nous en avons déjà parlé précédemment lors de l'examen d'amendements, et nous en reparlerons dans un instant. Il faut également agir sur le volet curatif, en améliorant les conditions de prise en charge de celles et de ceux qui développent des pathologies liées à cette exposition. On ne peut l'ignorer, certains utilisateurs ont été exposés à ces produits pendant une dizaine d'années, à une époque où le risque sanitaire était moins bien identifié, il faut le reconnaître. Lors d'une table ronde organisée par notre commission sur ce sujet, en janvier 2016, réunissant l'ensemble des parties prenantes, tous les acteurs convergeaient vers la nécessité d'assurer une meilleure indemnisation des victimes de ces produits, au premier rang desquels les agriculteurs. Par ailleurs, nous connaissons les limites du tableau des maladies professionnelles, qui a certes connu des évolutions, mais qui ne répond pas pleinement à la diversité des difficultés rencontrées par les malades. Vous avez parlé de l'amiante.

Je salue l'initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, engagée sur ce sujet depuis de nombreuses années, et je remercie Mme la rapporteur de la commission des affaires économiques pour l'avis favorable donné à cet amendement de compromis.

alors que, avec les produits phytosanitaires, le spectre est beaucoup plus large : comment apporter la preuve réelle que ce sont les produits phytosanitaires qui ont engendré la pathologie ? Voilà où est toute la difficulté. C'est pourquoi nous voulons

que les maladies liées aux produits phytosanitaires ne sont pas spécifiques. En clair, une même maladie peut être liée à une exposition à des produits phytosanitaires,

le tableau des maladies professionnelles. C'est la voie que nous avons choisie pour agir. La parole est à M. Joël Labbé,

Le scrutin est ouvert.

pour lesquelles les traitements traditionnels diffusés « à la main » ont tendance à exposer fortement les professionnels aux pesticides et, surtout, à déverser parfois trop de pesticides sur les pentes à accès difficile.

permettrait l'utilisation à moindre dose de ces produits de traitement. L'utilisation d'appareils volant très bas évite la dispersion du produit à laquelle donnait lieu l'épandage par hélicoptère. Elle renforce la sécurité des travailleurs. L'article 14 n'ouvre pas la porte à un nouvel épandage aérien démesuré et généralisé. Il s'agit d'une expérimentation, encadrée dans le temps, sur des surfaces en particulier, avec des pentes supérieures à 30 %, et qui fera l'objet d'une évaluation de l'ANSES. Pour toutes ces raisons, notre groupe souhaite le maintien de cet article dans sa rédaction actuelle. Je profite de cette occasion pour préciser que les drones ne sont pas uniquement utilisés pour l'épandage ; ils permettent également aux agriculteurs d'étudier l'évolution des cultures : ces derniers se servent des images de leurs champs pour optimiser l'usage des traitements et gérer au mieux les apports hydriques. on possède un drone, encore faut-il pouvoir l'utiliser. Or la réglementation en vigueur me paraît complexe et contraignante, peu adaptée à l'usage que peuvent en faire les agriculteurs.

En effet, au milieu d'une série d'articles visant à restreindre l'usage des intrants chimiques en agriculture, il autorise l'expérimentation d'épandage par drone. Il paraît que cela permettrait un épandage plus précis et moins dispendieux. Le bon sens paysan nous invite plutôt à penser que le moindre coup de vent capricieux viendra répandre les produits à côté de leur cible, abîmant un peu plus la biodiversité. C'est pour cette raison évidente que l'épandage aérien est interdit et qu'il doit le rester. N'ouvrons surtout pas la boîte de Pandore dans ce texte ! De surcroît, cette disposition ouvre la possibilité d'épandre des pesticides dans des zones jusque-là inaccessibles aux machines et aux pulvérisateurs. Nous pensons, notamment, aux cultures de moyenne montagne, que mon collègue Guillaume Gontard, qui siège à mes côtés, connaît bien. Ces terres jusqu'à présent préservées de pesticides seront désormais à la portée des intrants chimiques nous ne pouvons pas y voir un progrès. Enfin, la mécanisation incessante de l'agriculture constitue une fuite avant, qui oblige les agriculteurs à s'endetter toujours davantage pour « moderniser » leur exploitation. Cela diminue d'autant plus leurs marges financières et les place dans une situation de dépendance à l'égard de l'industrie. Tout cela les maintient dans un cercle vicieux dont ils ne peuvent plus sortir. N'aggravons donc pas les choses avec une nouvelle invention hors de prix, qui n'améliorera pas la situation des agriculteurs, mais aggravera encore peu plus la dégradation de nos sols. La parole

L'épandage de pesticides par voie aérienne pose des problèmes de santé publique et d'environnement du fait de la dérive au vent des produits pulvérisés. Il s'agit d'une pratique inadaptée au contexte agricole français en raison du parcellaire et de la densité des cours d'eau et des habitations. Les épandages aériens sont aujourd'hui interdits pour ces raisons. Il convient de rester sur cette position et d'éviter par cette expérimentation de rouvrir la porte aux épandages aériens. Il est certes proposé ici une simple expérimentation, mais ne mettons pas un pied dans la porte, qui est une porte de sortie. Nous devons, plutôt que revenir en arrière, promouvoir les alternatives qui existent. Par ailleurs, la législation actuelle et celle qui est proposée ne permettent pas d'assurer un contrôle efficace de l'usage des drones et, donc, une protection de la santé des riverains. Par conséquent, l'amendement vise à supprimer cette possibilité d'expérimentation. Pourquoi vouloir faire des drones le futur de l'agriculture ? J'ai lu voilà peu ? J'ai lu voilà peu de temps dans la presse que les super-fabricants de drones avaient réussi à imaginer des micro-drones à même de remplacer les abeilles pour assurer la pollinisation. C'est ce qu'on appelle l'« agriculture intelligente ». Si c'est ça l'intelligence,

dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien, qui se justifie avant tout, mes chers collègues, par la dangerosité pour les agriculteurs qui pulvérisent manuellement sur des surfaces présentant des pentes supérieures à 30 %.

des risques et la réduction de la dérive, grâce à des vols précis et de faible hauteur. Nous avons souhaité faire une expérimentation dans des conditions précises, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé, puis faire évaluer les résultats par l'ANSES. Cela permettra d'établir si ce mode d'application peut apporter les bénéfices attendus dans les conditions requises pour la santé et l'environnement.

L'amendement vise à mieux encadrer cette utilisation en raison des risques pour la santé publique ou l'environnement, en permettant une expérimentation exclusivement avec des produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification de très haut niveau d'exigence environnementale. environnementale. Il s'inscrit pleinement dans la perspective française de réduction d'usage des produits phytopharmaceutiques, notamment au travers du plan Écophyto II.

Je tiens ici à faire un rappel de l'évolution de cet article. Introduit en commission à l'Assemblée nationale, il n'autorisait initialement la pulvérisation aérienne que pour les vignes présentant des pentes supérieures à 30 %. 30 %. En séance publique, face aux critiques fortes émanant de plusieurs groupes politiques, il a été étendu à toutes les cultures présentant des pentes supérieures à 30 %. Il y était toutefois précisé que seuls les produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification haute pouvaient être épandus. Au Sénat, en commission, la rapporteur a étendu cette possibilité à tous les produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant cette possibilité sur toutes les cultures. Le texte que nous examinons aujourd'hui constitue donc clairement

Le rappel de l'évolution de cet article en est une illustration : au départ circonscrite, cette interdiction est désormais généralisée à l'ensemble du territoire avec des produits conventionnels. Si nous votons le texte en l'état, un autre viendra encore ouvrir le champ des dérogations et nous en reviendrons au point de départ. De plus, pour ce qui est de la pente de 30 %, nous restons très dubitatifs sur les moyens dont nous disposerons pour vérifier que les conditions sont réellement remplies. Selon moi, nous ouvrons ici la voie à toutes les dérives. C'est pourquoi je vous propose d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale : une dérogation pour les surfaces présentant une pente supérieure à 30 % uniquement pour les produits autorisés en agriculture biologique ou présentant une certification HVE

quel que soit le produit. Il est possible de prévoir que l'arrêté interministériel qui définira les conditions d'expérimentation restreigne celles-ci à certains produits, mais selon des caractéristiques autres que leur origine naturelle.

pas pour l'épandage de produits phytosanitaires, mais pour d'autres objets, par les agriculteurs dans des zones à faible risque. L'agriculture utilise déjà- ce chiffre est d'ailleurs stupéfiant -la moitié des 20 000 drones civils en service. Grâce aux images prises par leur capteur, ces drones volants donnent des indications agronomiques, sans qu'il soit besoin d'effectuer de prélèvements. En survolant une parcelle, un drone enregistre une multitude d'images géoréférencées avec une précision centimétrique. C'est sa faible altitude- 150 mètres -, par rapport à celle d'un satellite, qui lui permet cette précision. Plus de 10 000 hectares ont été survolés en 2016. Dans mon département, la Somme, sont même devenus un outil du quotidien depuis que la chambre d'agriculture s'est équipée en 2013 et les met à disposition des agriculteurs. La chambre d'agriculture poursuit ses expérimentations pour affiner la modulation

Ces formalités rendent quasi obligatoire le passage par un prestataire, ce qui limite considérablement le développement de ces outils, qui sont pourtant facteur de durabilité de notre agriculture. permettrait donc, s'il était adopté, comme je l'espère, de libérer l'usage des drones agricoles en respectant des conditions d'emploi strictes pour éviter tout incident avec l'aviation habitée. Les inquiétudes qui ont pu s'exprimer en commission trouvent une réponse, premièrement, dans la limitation de la masse- 800 grammes au lieu de 2 kilos -, afin d'entrer dans le champ d'application de la loi et, deuxièmement, dans la finalité économique et environnementale de l'usage des drones dans le milieu agricole. Cela explique la nécessité d'une réglementation différente pour les agriculteurs. Quel

En outre, l'amendement prévoit des dérogations spécifiques à la formation pour le survol dans les zones non peuplées qui ne sont pas prévues par la loi de 2016, qui n'est d'ailleurs pas encore en vigueur. Laissons-nous le temps d'apprécier l'efficacité de cette loi. L'avis est donc défavorable. Quel est

pour interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement habitées. Il répond à un enjeu d'exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Ces riverains sont impuissants face aux pratiques des agriculteurs, alors que ceux-ci épandent parfois des pesticides jusque sous leurs fenêtres. Ils réclament pourtant, à juste titre, une protection. Certaines études tendent à établir un lien entre l'exposition non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et des pathologies chroniques. Par exemple, le rapport de l'INSERM de 2013 intitulé atteste de leur impact non seulement sur les agriculteurs, mais aussi sur les riverains des zones cultivées. Il évoque ainsi plusieurs études montrant une augmentation du risque de malformations congénitales, de tumeurs cérébrales et de leucémies chez les enfants des femmes vivant au voisinage d'une zone agricole. Ces effets liés à une exposition au long cours sont parfois très difficiles à établir. Bien des riverains témoignent de troubles de santé manifestes : irritations oculaires, problèmes respiratoires, malaises. Des mesures sont prévues pour protéger, par exemple, les écoles, mais les enfants peuvent aussi être exposés chez eux, dans leur habitation. Pourquoi ne pas prévoir la possibilité de prendre des mesures en ce sens ? Certes, parfois, des solutions locales sont trouvées par le dialogue entre riverains et agriculteurs, ce qui est la meilleure des solutions, mais pas dans tous les cas. L'intervention de l'autorité administrative est donc essentielle pour trouver des solutions locales et protectrices. Il s'agit là d'un amendement très modéré. L'autorité administrative n'est pas tenue de prendre des mesures : elle peut les prendre, par exemple, seulement pour certaines catégories de produits. Je pense notamment- et je n'ai pas fini d'en parler -aux pesticides cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ces mesures sont d'ailleurs recommandées dans le cadre du règlement CE n° 1107/2009 et de la directive-cadre sur l'utilisation des pesticides.

Il vise à autoriser l'autorité administrative compétente à prendre des mesures pour restreindre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement habitées. Il s'agit ici de prendre les dispositions adéquates pour protéger les riverains d'exploitations agricoles, ce qui est une demande très souvent formulée par les riverains de ces exploitations qui subissent des épandages de certains produits à quelques mètres de leur habitation, avec les conséquences que cela peut avoir pour la santé des personnes concernées. Je précise qu'il ne s'agit en aucun cas d'interdire les épandages, car ce n'est pas l'objet de notre texte. Il s'agit de renforcer les pouvoirs du préfet, qui lui permettent, lorsque la situation l'exigera, de prendre des dispositions adéquates pour protéger nos concitoyens. Les réponses à cette question sensible ne peuvent passer que par la discussion, l'échange, la concertation, le respect de tous. Je connais ce problème dans mon département, qui est très viticole. J'ai aussi bien connu cette problématique en Corrèze avec les pomiculteurs : les choses ont pu se régler grâce à la mise en place d'une charte. Je sais quelles propositions fera M.

Cet amendement vise à permettre aux préfets de définir des mesures d'interdiction ou d'encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des mesures de protection adaptées dans les zones attenantes aux bâtiments habités. Un rapport d'inspection de décembre 2017 avait préconisé une telle mesure pour réduire l'exposition de la population aux produits phytopharmaceutiques, notamment celle des femmes enceintes et des enfants en bas âge, qui sont directement affectés, comme l'INSERM l'avait souligné dans son rapport de 2013. Pas plus tard que lundi dernier, l'ANSES, l'INERIS et les associations de surveillance de la qualité de l'air ont annoncé une nouvelle campagne sur la mesure des pesticides dans l'air. Il s'agit donc d'un sujet sur lequel les pouvoirs publics convergent pour mieux protéger la population, et nous devons y contribuer. du développement durable prévoit de faire précéder ces mesures d'une consultation des riverains, des exploitants agricoles et des collectivités territoriales concernées, afin de rechercher des solutions partenariales avec des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, cette rédaction fait référence à des mesures de protection adaptées, par analogie avec le régime applicable à proximité des établissements accueillant un public vulnérable. Il s'agit de souligner que cette décision sera prise lorsque les circonstances locales le justifieront dûment et que les mesures pourront prendre différentes formes : plantations de haies, équipements utilisés au moment du traitement ... Au final, l'amendement de notre commission prévoit un dispositif clair et équilibré pour renforcer la prévention des risques et répondre à une attente forte, clairement exprimée lors des États généraux de l'alimentation.

à la concertation, qui est nécessaire sur toutes les questions relatives aux traitements. Les chartes existent d'ores et déjà en viticulture. Il convient d'en promouvoir le développement. Je veux appeler votre attention sur le fait qu'il n'y a plus

De plus, les maires, à défaut les préfets, disposent d'un pouvoir de police générale sur leur territoire en cas de risque pour la salubrité publique. Ils peuvent déjà prendre ces dispositions et les adapter le plus finement à la réalité du terrain. Nous mesurons à quel point cette adaptation est importante.

Or les amendements présentés aujourd'hui ouvrent la porte à une interdiction automatique par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. C'est une remise en cause du pouvoir d'appréciation du maire et une véritable restriction de la libre administration des collectivités territoriales. Le maire est l'autorité la plus à même de réaliser des médiations entre les riverains et les agriculteurs sur ces sujets et d'identifier le plus précisément possible à la fois les parcelles concernées et le dispositif à mettre en place. Prévoir de telles possibilités dans la loi reviendrait à limiter ces marges de manoeuvre, d'autant que ces sujets sont susceptibles de trouver des solutions dans le cadre des plans locaux d'urbanisme.

l'enjeu était la réduction de près de 4 millions d'hectares de surface agricole utile, soit 14 % de la surface agricole dite utile. La commission insiste sur le mécanisme des chartes entre riverains et producteurs sous l'égide du maire. Ces initiatives locales ont fait d'ores et déjà la preuve de leur efficacité et elles sont aujourd'hui nécessaires pour prendre des mesures réellement adaptées aux réalités du terrain.

Nous avons pris un certain nombre de mesures pour les agriculteurs, notamment pour les protéger, nous l'avons vu tout à l'heure : l'amendement de Mme Bonnefoy a été adopté à l'unanimité, et j'en comprends parfaitement la raison. Reste que nous avons besoin aussi

que l'on empêche les agriculteurs et les producteurs de travailler dans de bonnes conditions et de valoriser leur terre et leur territoire.

dizaines de microns et qui dérivent pas mal. On peut très bien traiter à des dizaines ou à des centaines de mètres des habitations et ressentir les produits qui sont utilisés.

prenez-vous-en à ceux qui fabriquent ces produits-là ! Prenez-vous-en à ceux qui autorisent la commercialisation de ces produits ! Arrêtez de taper sur les agriculteurs

de projeter des molécules sur les plantes à raison de 2 462 points d'impact recto verso sur une feuille grâce à des buses de pulvérisation, grâce à des adjuvants et à des buses anti-dérives, qui permettent de localiser le produit là où il faut, quand il faut.

de construire du dialogue territorial et de faire confiance aux acteurs du territoire. Pour ma part, je pense qu'en ce 2 juillet, alors que nous étions tous hier sur nos routes départementales et que ce matin nous avons tous mis à jour nos applications GPS,

Monsieur le ministre, ce sont des zones de non-traitement ou des zones de non-agriculture ou de non-vigne que vous voulez mettre en place ! D'un côté, quand vous parlez à la profession, vous lui proposez des espaces de négociations et de discussions dans le plan de filière. La profession, notamment viticole, a pris des engagements très forts qu'elle va mettre ou qu'elle met déjà en oeuvre : plantations de haies, remembrements de parcelles, essais de cépages résistants. D'un autre côté, une fois dans l'hémicycle- loin des yeux, loin du coeur -, vous proposez un amendement customisé ... Ah ! ... pour obtenir le sésame du Sénat.

vous allez même englober l'agriculture bio. C'est désespérant ! L'État ne doit pas faire dans le cosmétique : il doit prendre ses responsabilités. Vous devez demander à l'ANSES de définir au cas par cas les précautions à prendre pour les riverains, dans le cadre des autorisations de mise sur le marché, ainsi que l'Europe l'impose. Si l'ANSES ne veut pas le faire, car elle estime que le produit présente un risque, alors elle doit retirer l'homologation du produit. Monsieur le ministre, respectez vos engagements et votre promesse de discussions dans le plan de filière. Cessez de faire peur à la population !

qui se propageront aux parcelles voisines. Il faudra donc utiliser encore plus de produits pour enrayer les épidémies. Et il y en a ! Parfois, c'est l'oïdium, parfois c'est le mildiou. Si l'on ne traite pas tout de suite les endroits où se déclare la maladie, c'est l'ensemble du vignoble qui est touché.

par caractéristiques géologiques, la vigne appellation champagne pousse sur ces pentes-là. Les habitations se sont développées au coeur de ces cultures

est un engagement mutuel consenti entre plusieurs personnes ou groupes de personnes, en l'occurrence entre des agriculteurs et des riverains. C'est

et à celles des riverains. Les chartes sont adoptées localement, de manière à fixer les conditions de traitement les plus favorables au cas par cas. Il faut prendre en compte un certain nombre de principes,

est ainsi libellé : La parole est à Mme Angèle Préville. Le 5 avril dernier, 217 élèves des écoles de plusieurs communes des Deux-Sèvres ont été incommodés par l'épandage de produits phytosanitaires sur le site même où ils étaient rassemblés à l'occasion d'une course d'orientation organisée dans le cadre d'une sortie scolaire.

Il convient que la législation prenne en considération la nécessaire protection des enfants, non seulement dans les crèches et dans les écoles, mais aussi dans tout lieu où ils peuvent être amenés à se trouver rassemblés. Dans ce cas, l'autorité administrative doit pouvoir déterminer un périmètre de zone de non-traitement temporaire.

relève des pouvoirs de police générale du maire et du préfet, la salubrité publique étant en jeu, dans la mesure, ma chère collègue, où ils ont bien été informés préalablement d'un risque occasionnel. J'émets, au nom de

tenu de cela et du caractère volatile des pesticides, leur épandage est déjà interdit près des écoles et des hôpitaux, pour protéger les populations les plus fragiles. J'ai entendu tout à l'heure affirmer que les cultures bio pouvaient contaminer les autres : un comble ! Il nous semble important,, de protéger les cultures biologiques de la contamination par les pesticides. Les consommateurs se tournent vers les produits biologiques justement pour éviter ceux-ci. Ce label est garanti par l'Union européenne. C'est une boussole pour nombre de nos concitoyens désireux de consommer plus sainement. Nous ne pouvons pas, en toute honnêteté, imposer une réglementation exigeante aux agriculteurs pour l'obtention de ce label et fermer les yeux sur la contamination de leurs champs par les pesticides utilisés leurs voisins. C'est tromper le consommateur ! Enfin, cette mesure vise à protéger les agriculteurs qui font de gros efforts pour acquérir le label bio. De plus en plus, les agriculteurs se tournent vers la production biologique. Ils méritent d'être respectés dans leur choix et donc d'être assurés d'une protection contre la contamination par les pesticides. Quel

Cet amendement de repli est plus minimaliste encore que le précédent. Il vise à garantir l'information des riverains. J'ai été interpellé localement par un collectif de riverains qui m'a demandé de voir s'il était possible d'instaurer,

d'habitations, les riverains sont en droit de savoir qu'une parcelle est en cours de traitement ou qu'elle vient d'être traitée et qu'il est donc dangereux d'y pénétrer. Les parcelles agricoles relèvent certes de la propriété privée, mais des enfants peuvent malgré tout, à un moment ou à un autre, décider d'y entrer et s'exposer ainsi, dans le cas où il vient d'être procédé à un épandage, à des substances dangereuses.

Cet amendement vise donc à mettre en place une signalisation claire pour avertir le public. Puisqu'il y a refus de prendre des mesures réellement contraignantes, ce que je déplore, garantissons au moins la transparence de l'information.

Quelle est la responsabilité du législateur, si ce n'est, justement, de s'éloigner des considérations économiques pour s'attacher à des considérations de sécurité ? Dieu sait si la sécurité alimentaire est au coeur de nos débats ! C'est la raison pour laquelle je pense profondément, monsieur le ministre, que vous ne prendriez aucun risque à approuver cet amendement, qui concerne la protection des consommateurs et n'est en rien motivé par des considérations de compétition ou de compétitivité internationale. C'est le consommateur qui est notre préoccupation, et c'est votre devoir de le défendre

l'essentiel, les points critiques révélés par l'ANSES dans son étude réalisée pour servir de base à l'arrêté fixant ces dérogations relèvent de freins économico-commerciaux, et non de réelles impasses techniques. Ces freins peuvent être levés non par des dérogations à l'interdiction des néonicotinoïdes, mais par des mesures d'accompagnement et de soutien. Rappelons par ailleurs que des études réalisées sur plusieurs grandes cultures ont fait valoir que l'utilisation des néonicotinoïdes n'a pas permis

Depuis l'adoption de l'interdiction en 2016, les études sur la toxicité de ces pesticides n'ont cessé de s'accumuler. Par exemple, une étude allemande de 2017 révèle que les populations d'insectes volants ont diminué de 80 % en De même, une étude conjointe du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS a démontré que les populations d'oiseaux diminuaient « à une vitesse vertigineuse Ces deux études ont montré la responsabilité des néonicotinoïdes dans ces phénomènes. L'urgence de la situation justifie de n'accorder aucune dérogation à cette interdiction.

Cet article permet de consolider l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, en évitant son contournement par le recours à des produits présentant des modes d'action identiques.

afin de garantir que ces mesures réglementaires se fonderont sur des données scientifiques, en particulier pour la définition de la notion de mode d'action. Il y a des produits de même mode d'action dont les métabolites sont très peu toxiques, qui sont peu rémanents dans le milieu environnant et qui peuvent donc être considérés comme de très bons produits et de bonnes solutions alternatives.

à M. le ministre. Il s'agit de rétablir l'article 14 , qui concerne l'extension de l'interdiction des néonicotinoïdes aux substances présentant un mode d'action identique. L'Europe a décidé, le 27 avril 2018, d'interdire le traitement des cultures en plein champ utilisant trois des substances néonicotinoïdes à compter de la fin de 2018. Cette décision, qui concerne plus de 76 % de la des quantités et intervient six ans après les premières mesures nationales, vient confirmer la position française sur la nécessité de mieux protéger les insectes pollinisateurs. Il convient désormais d'étendre le champ de l'interdiction aux substances chimiques qui, si elles ne sont pas classées spécifiquement comme néonicotinoïdes, ont des modes d'action identiques, car c'est le mode d'action qui est incriminé, notamment en matière d'impact sur les pollinisateurs, dont on connaît la situation préoccupante aujourd'hui. Un décret précisera la liste des modes d'action à prendre en compte pour la mise en oeuvre de la disposition.

Nous proposons donc d'étendre cette interdiction à des substances dont les modes d'action sont identiques à ceux-ci. L'objectif est d'éviter tout contournement de la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016. En effet, de nouvelles substances, telles que le sulfoxaflor et la flupyradifurone, ont été depuis créées. Le débat sur leur appartenance ou non à la famille des néonicotinoïdes n'est pas encore tranché. Or, rappelons-le, sont désastreux sur les pollinisateurs, notamment sur les abeilles. Ces substances agissent en effet sur leur système nerveux central, leur faisant par exemple perdre le chemin de leur ruche. C'est donc bien leur mode d'action qui présente un danger. Ces substances mettent en question la préservation des espèces, alors que les populations d'insectes volants connaissent un déclin considérable. Rappelons que l'action des pollinisateurs est essentielle pour les écosystèmes et pour nos cultures, puisque les trois quarts de

nous devons nous prémunir contre les dangers que peuvent présenter de nouvelles substances, qu'elles soient classées comme néonicotinoïdes ou non, pour les pollinisateurs.

Il vise également à rétablir l'extension du champ d'application de l'interdiction des néonicotinoïdes aux substances ayant un mode d'action similaire, telle qu'elle a été proposée par l'Assemblée nationale. Ces substances sont des neurotoxiques, qui affectent le système nerveux central des insectes,

Cette extension est indispensable au regard de la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les apiculteurs et l'ensemble de la biodiversité. Ces pesticides ayant le même mode d'action que les néonicotinoïdes, il est complètement justifié qu'ils soient eux aussi interdits pour protéger les pollinisateurs, notamment. C'est en effet le mode d'action systémique de ces pesticides qui représente un danger pour les abeilles. Vous le savez, la situation des pollinisateurs est catastrophique. Cette année, la mortalité dans certaines régions a été particulièrement importante. Les apiculteurs ont interpellé à de multiples reprises les pouvoirs publics sur leur situation, économiquement

n° 636 rectifié. Le 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de deux formulations commerciales à base de sulfoxaflor, un nouvel insecticide apparenté aux néonicotinoïdes. L'autorisation accordée ne respectait pas le principe de précaution. En effet, selon le tribunal, il n'existait pas de certitude quant à l'innocuité de ce produit. Par cet amendement, nous souhaitons apporter une réponse politique à cette situation. Nous entendons prendre nos responsabilités à l'égard de nos concitoyens, en les protégeant contre ces nouveaux pesticides. chers collègues, vous avez défendu en commission la filière apicole par l'amélioration de l'étiquetage du miel et nous soutenons cette mesure. Soutenez jusqu'au bout cette filière en interdisant complètement ces nouveaux pesticides tueurs d'abeilles.

nous devons nous donner les moyens de contrecarrer toute tentative de détournement de l'esprit de la loi. Nous proposons également, en cohérence avec l'interdiction actuelle des néonicotinoïdes, de prévoir que cette mesure entre en vigueur le 1 septembre 2018.

Ces dérogations, très peu nombreuses, sont accordées uniquement jusqu'au 1 juillet 2020 dans la mesure où il n'existe aucun substitut, chimique ou non. L'amendement

L'Europe a décidé, le 27 avril 2018, d'interdire le traitement des cultures en plein champ utilisant trois des substances néonicotinoïdes à compter de la fin de 2018. Cette décision, qui concerne plus de 76 de la population, intervient plus de six ans après les premières mesures nationales et vient confirmer le bien-fondé de la position française sur la nécessité de mieux protéger les insectes pollinisateurs.

maritimes. De sérieux doutes pèsent sur l'efficacité de l'alternative présentée par l'ANSES, car il n'existe aujourd'hui aucun traitement de substitution.

J'attends de vous, monsieur le ministre, un engagement ferme sur l'octroi d'une dérogation à l'utilisation de ces produits pour la filière betterave. Il y va de sa survie. Je vous demande, monsieur le ministre, d'être fidèle à vos déclarations de cet après-midi.

permettre de traiter les problèmes sans difficulté. Aucune dérogation à ce stade n'est possible pour un néonicotinoïde interdit depuis le 27 avril dans toute l'Europe

Le scrutin est ouvert.

Cet amendement vise à interdire la production, le stockage et la vente de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées à l'échelon européen. Il avait été adopté par la commission du développement durable à l'Assemblée nationale, avant d'être rejeté en séance par le Gouvernement, au motif qu'il tendrait à pénaliser notre industrie. Or nous estimons qu'il s'agit ici d'être cohérents avec nos politiques et nos engagements, tant nationaux qu'européens. Il me semble impensable de continuer à autoriser nos entreprises à exporter des substances que nous n'autorisons pas chez nous. La nocivité d'un produit ne s'arrête pas à nos frontières et elle ne diminue pas avec les kilomètres Nous devons être exemplaires si nous voulons être crédibles. Les considérations économiques qui ont conduit à la suppression de cet article à l'Assemblée nationale ne me convainquent pas. Il s'agit ici de santé publique mondiale, ainsi que d'éthique. Nous proposons cependant, afin de faciliter l'adoption de notre amendement, que cette interdiction prenne effet au 1 janvier 2020, pour laisser le temps aux entreprises concernées de s'organiser en conséquence.

de l'alimentation et des espaces ruraux, le Conseil général de l'environnement et du développement durable et l'Inspection générale des affaires sociales ont mis en avant le danger sanitaire que peuvent présenter certaines substances

dans ce domaine, comme nous l'avons été pour les néonicotinoïdes. Il est donc tout à fait logique, dans l'optique de la gestion des risques, de suivre cette évaluation des pesticides et de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires pouvant en contenir.

Ils s'appuient, comme cela a été dit, sur un rapport qui a identifié ces substances préoccupantes. Or ce rapport ne préconise nullement l'interdiction de ces substances actives par la loi. Il recommande, à juste titre, d'agir directement à l'échelon européen pour les faire interdire en demandant leur réévaluation. Je précise également que l'article 253-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toutes dispositions d'interdiction concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation ou la détention des produits

dispositions réglementaires européennes en vigueur, si cette évaluation fait apparaître des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'approbation européenne, ceux-ci seront transmis sans délai à la Commission européenne afin que soit engagée la révision de l'approbation. Si l'étude identifie des risques inacceptables,